La séance est reprise. L’ordre du jour appelle l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte. L’ordre du jour

Ces travaux ont conduit à l’adoption, en 2016, de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices. C’est dans ce cadre que la France a souhaité mettre à jour la convention franco luxembourgeoise du 1 avril 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Ainsi, les travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant leur activité au Luxembourg demeuraient soumis à l’impôt au Luxembourg, même lorsqu’ils travaillaient en dehors de ce pays, dans la limite d’un plafond de 29 jours de télétravail par an. Toutefois, si jamais ce seuil était dépassé, les dispositions de la convention étaient réputées ne pas s’appliquer et l’intégralité des jours de télétravail étaient alors imposés en France. Face à la pratique massive du télétravail constatée lors de la crise sanitaire, ce cadre juridique est cependant rapidement apparu obsolète. D’une part, nous sommes intervenus activement afin de neutraliser les effets fiscaux de ce recours massif au télétravail pendant cette période. L’épidémie ayant été considérée comme un cas de force majeure, des accords amiables ont été conclus avec les autorités luxembourgeoises pour instaurer un dispositif dérogatoire applicable à compter du 16 juillet 2020, puis reconduit jusqu’au 30 juin 2022. Pendant cette période, le dispositif prévoyait de ne pas prendre en compte les règles de calcul du forfait de télétravail inscrit dans la convention fiscale pendant la période délimitée précitée. D’autre part, dans la perspective d’un retour à la mise en œuvre normale des dispositions prévues dans la convention de 2018 et considérant l’essor du télétravail, le plafond de 29 jours est rapidement apparu obsolète pour ceux des 122 000 travailleurs transfrontaliers français concernés par le télétravail.

L’avenant à la convention fiscale signé le 7 novembre 2022, soumis à votre approbation, entérine cette décision. Plus précisément, cet accord prévoit que les jours de télétravail effectués dans la limite du plafond de 34 jours seront imposés comme s’ils avaient été effectués au poste de travail habituel dans l’État de situation de l’employeur. En revanche, au delà de cette limite, la totalité des jours télétravaillés sera imposée dans l’État où est physiquement exercée l’activité professionnelle. Les dispositions de cet avenant s’appliquent pour les revenus perçus à compter du 1 janvier 2023. Le relèvement du seuil de 29 à 34 jours reflète la réalité de l’emploi des Français travaillant au Luxembourg aujourd’hui et devrait avoir pour effet d’encourager cette nouvelle modalité d’exercice de l’activité professionnelle. La mesure devrait contribuer à améliorer la qualité de vie des travailleurs frontaliers en leur permettant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. De même, l’impact écologique du développement du télétravail n’est pas négligeable, puisqu’il conduit à une baisse de l’affluence sur les axes routiers et dans les transports en commun. En outre, afin de répondre à une demande du Luxembourg motivée par l’inégalité de traitement existante entre les salariés du secteur du secteur privé et les agents de la fonction publique, l’avenant étend le bénéfice du forfait de télétravail de 34 jours par an aux agents de la fonction publique. L’augmentation du seuil de 29 à 34 jours de télétravail illustre notre volonté commune de dynamiser la relation bilatérale entre la France et le Luxembourg en prévoyant une règle d’imposition claire qui réponde à une attente de nos compatriotes exerçant une activité professionnelle frontalière. Telles sont, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu’appelle l’avenant à la convention entre la France et le Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des finances a examiné et adopté ce projet de loi qui vise à approuver l’entrée en vigueur d’un avenant à la convention fiscale bilatérale entre la France et le Luxembourg. En application de l’article 53 de la Constitution, il appartient en effet au Parlement d’approuver ou de ratifier un certain nombre d’accords internationaux, dont font partie les conventions fiscales. Dans ce cadre, le Sénat est la première chambre saisie du présent projet de loi, qui comporte un article unique autorisant l’approbation de l’avenant du 7 novembre 2022 à la convention fiscale bilatérale du 20 mars 2018 entre la France et le Grand Duché de Luxembourg. Dans un premier temps, et préalablement à l’exposé du contenu de cet avenant, il me paraît opportun de rappeler les évolutions récentes de notre relation fiscale avec le Luxembourg. La France et le Luxembourg ont signé le 20 mars 2018 une nouvelle convention venant remplacer celle de 1958 qui régissait jusqu’alors nos relations en matière fiscale. La modernisation des relations bilatérales était attendue et nécessaire, notamment pour tenir compte des avancées en la matière de l’OCDE. Par conséquent, la convention intègre les derniers standards de l’OCDE, notamment une définition modernisée de la résidence fiscale et de la notion d’établissement stable, qu’une clause générale anti abus. Parmi les concessions obtenues par le Luxembourg au cours des négociations de la convention de 2018 figure un régime spécifique d’imposition du télétravail des transfrontaliers. Compte tenu de sa superficie et de sa situation géographique, le Luxembourg est en effet particulièrement dépendant de la main d’œuvre transfrontalière pour faire fonctionner son économie et ses services publics.

les deux ! – travaillent au Luxembourg, les deux premiers départements de résidence de ces transfrontaliers étant la Moselle et la Meurthe et Moselle. Le protocole annexé à la convention de 2018 prévoit ainsi un forfait de télétravail de 29 jours au cours duquel le contribuable est réputé travailler dans l’autre État. Concrètement, un Français qui travaille au Luxembourg est, en principe, imposé au Luxembourg. Lorsqu’il télétravaille en France jusqu’à 29 jours, il est réputé exercer son emploi au Luxembourg et continue donc d’être imposé dans ce pays. Je précise que cette clause est de nature fiscale et n’empêche en rien de télétravailler au delà de 29 jours. Simplement, en cas de dépassement du seuil, l’activité est imposée dans l’État de résidence dès le premier jour de télétravail. Les règles d’application de la convention ont été précisées dans un accord amiable du 16 juillet 2020, qui fixe notamment la méthode de décompte des jours de télétravail. Si ce régime permet de simplifier la situation des transfrontaliers, il conduit à une perte fiscale pour la France, estimée entre 30 millions d’euros et 60 millions d’euros annuels par la direction de la législation fiscale. La France renonce en effet à un droit à imposer les activités en télétravail en deçà de 29 jours. Cette perte fiscale peut être en partie compensée par les recettes de TVA induites par les dépenses en France des télétravailleurs. En dépit de ce manque à gagner fiscal, au sortir de la crise sanitaire, au cours de laquelle le télétravail s’est banalisé, les gouvernements français et luxembourgeois se sont accordés pour étendre le forfait de télétravail. J’en viens donc au second point de mon intervention, qui aborde plus en détail les stipulations de cet avenant. S’il est vrai que son contenu et sa portée sont relativement limités, son entrée en vigueur est attendue, à la fois par les travailleurs transfrontaliers et par notre partenaire luxembourgeois. Premièrement, l’avenant augmente donc la durée du forfait de télétravail de 29 à à 34 jours. Désormais, le seuil de 34 jours conditionne le régime d’imposition des contribuables en télétravail. Ce seuil de 34 jours correspond à une demande des autorités luxembourgeoises. Il est cohérent avec la renégociation récente par le Grand Duché de ses conventions avec la Belgique et l’Allemagne afin de prévoir des seuils similaires de télétravail à 34 jours. Cette renégociation d’ensemble permet de placer les travailleurs transfrontaliers sur un pied d’égalité, quel que soit leur pays d’origine. Deuxièmement, l’article 2 de l’avenant étend le bénéfice du forfait de télétravail à certains contribuables percevant des rémunérations publiques. La technicité de cette clause mérite de s’y attarder un instant. La convention de 2018 prévoit deux hypothèses d’imposition pour les contribuables percevant des rémunérations publiques. Le principe général est que ces rémunérations sont imposées dans l’État de source. Concrètement, un Français travaillant au Luxembourg pour l’ambassade de France est imposé en France. Par exception, la convention précise que les rémunérations publiques sont imposées dans l’État d’exercice de l’activité lorsque le contribuable est résident de cet État et dispose de sa seule nationalité. Lorsqu’un Luxembourgeois travaille au Luxembourg pour l’ambassade de France, il est imposé au Luxembourg. Or le télétravail peut faire basculer un contribuable d’une hypothèse à l’autre. Un Français qui travaille pour la ville de Luxembourg est imposé au Luxembourg en présentiel et en France en télétravail. Pour remédier à cette situation, l’avenant permet de prévoir qu’en deçà du seuil de 34 jours de télétravail les revenus sont imposés dans l’État de source. Cette stipulation permet d’aligner le régime des personnes employées dans le secteur public sur le régime des personnes employées dans le secteur privé. Troisièmement, l’avenant prévoit une clause de revoyure à la fin de 2024, qui permettra aux parties à la convention d’examiner l’application de ces nouvelles règles. Cet examen devrait permettre d’envisager un nouveau régime d’imposition du télétravail transfrontalier. En effet, les règles actuelles apparaissent comme un cadre provisoire. En l’état du droit, il s’agit d’un compromis équilibré, qui permet de concilier la simplification de la situation administrative des travailleurs transfrontaliers et la protection des intérêts du Trésor public. Cependant, je pense qu’il serait opportun, à l’avenir, de rehausser le forfait de télétravail, auquel les travailleurs transfrontaliers sont très favorables, et, en même temps, d’envisager une meilleure répartition des recettes fiscales entre

travail, soit deux jours par semaine, au cours duquel s’applique le principe d’imposition dans l’État d’exercice de l’activité. En contrepartie, l’État qui dispose du droit d’imposer reverse une compensation fiscale à l’État de résidence. Dans l’attente de cette renégociation, l’entrée en vigueur de l’avenant soumis à notre approbation me paraît nécessaire pour simplifier le régime d’imposition des travailleurs transfrontaliers.

Le télétravail, autrefois considéré comme un privilège ou une exception, s’est imposé comme un élément central de notre quotidien professionnel. Cette évolution rapide a démontré que le travail à distance n’était pas uniquement viable, mais qu’il apportait également de nombreux bienfaits tant pour les employés que pour les entreprises. Son adoption massive et sa pérennisation posent toutefois de nouvelles questions, notamment en matière d’organisation du travail et de fiscalité transfrontalière. C’est dans ce contexte que la modification de la convention fiscale avec le Luxembourg prend tout son sens. En augmentant le nombre de jours de télétravail pendant lesquels les travailleurs résidents l’un des deux États et employés par l’autre ne sont pas imposés par leur État de résidence, faisant passer ce seuil de 29 à 34 jours, nous reconnaissons les changements intervenus dans notre façon de travailler. envoyons un signal à nos 120 000 compatriotes travaillant au Luxembourg, ainsi qu’à leurs employeurs, en les assurant que le cadre législatif évolue en phase avec les réalités du monde professionnel.

En étendant cette flexibilité fiscale aux fonctionnaires transfrontaliers, nous permettons à tous les travailleurs de bénéficier des mêmes droits et opportunités dans le cadre de leur activité professionnelle. En outre, en prévoyant une nouvelle discussion des autorités des États d’ici à la fin de 2024, l’avenant consacre une démarche d’évaluation et d’ajustement continus

Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI soutiendra cet avenant, qui représente une avancée vers un cadre de travail plus moderne et adaptable,

la convention fiscale ne répond pas à cette ambition, car elle ne gratifie le contribuable que de moins d’une journée par semaine de travail à distance. Elle ne règle pas non plus l’enjeu du partage de la ressource fiscale ou celui de la nécessaire simplification administrative. La question

Les Luxembourgeois eux mêmes, parce qu’ils subissent l’envolée des prix de l’immobilier dans leur territoire, sont nombreux à élire domicile dans les communes frontalières, ce qui aggrave encore l’engorgement du trafic L’attractivité économique du Grand Duché n’en finit pas d’attirer les frontaliers, qui, en retour, sont indispensables au maintien, au développement et à la croissance de l’économie luxembourgeoise. Si le Luxembourg veut en effet maintenir son niveau de développement économique actuel, on estime qu’il lui faudra plus de 9 000 nouveaux travailleurs étrangers par an d’imaginer que cela pose un problème en matière non seulement de mobilité vers le Luxembourg, mais aussi de locaux de travail disponibles dans ce petit pays. On l’aura compris, le recours au télétravail est indispensable tant pour les travailleurs français que pour les employeurs luxembourgeois, et il le sera toujours plus à l’avenir. donc fixer ce seuil à 34 jours, alors que l’on pourrait raisonnablement aspirer à une cinquantaine de jours télétravaillés ? Le choix de ce nombre vient du Luxembourg, qui travaille, paraît il, à la cohérence de sa politique conventionnelle avec ses voisins.

Je termine en plaidant en faveur d’une plus grande coopération et harmonisation à l’échelle de la Grande Région. Nous devons renforcer l’intégration politique, ainsi que la collaboration économique et fiscale à une échelle globale. Si l’on veut vraiment traiter sur un pied d’égalité toutes les entités devenues interdépendantes, celles ci doivent avoir la volonté politique de s’accorder et de décider en commun, et non plus au cas par cas, à la faveur de multiples traités bilatéraux aux conditions variables. La parole est

Si les effets du télétravail au sein des entreprises sont encore incertains, j’estime que cet avenant est bénéfique pour les travailleurs

vie de ces travailleurs. Monsieur le ministre, j’appelle votre attention sur le fait qu’il s’agit là de la deuxième modification de la convention depuis son entrée en vigueur en 2019. en vigueur en 2019. Nous avons déjà examiné en 2020 un avenant revenant sur les modalités d’imposition des revenus d’emploi des travailleurs transfrontaliers. Par ailleurs, le présent avenant comporte une clause de revoyure, qui laisse entrevoir une nouvelle modification au cours des prochains mois. Ces modifications successives révèlent, selon moi, un véritable problème de méthode dans la conduite de nos relations transfrontalières avec le Luxembourg. Tout les modalités actuelles de négociation des conventions fiscales ne prennent pas assez en compte les spécificités de notre relation bilatérale avec le Luxembourg.

il importe de se projeter au delà des stipulations techniques afin d’anticiper les modalités et, parfois, les difficultés de mise en œuvre à l’échelon local. local. Monsieur le ministre, nous devons faire ce travail au niveau politique, en associant l’ensemble des acteurs de la coopération transfrontalière. Ce travail d’anticipation dépasse, à mon sens, le domaine exclusivement fiscal. La coopération transfrontalière englobe les domaines de la santé, de l’emploi, des transports, de la sécurité, et bien d’autres que nous devons cesser d’appréhender un par un et de manière purement technique. Ces sujets ne sont pas indépendants les uns des autres.

le cadre de notre coopération transfrontalière me paraît pour le moins perfectible. À l’échelon des deux états comme à celui des collectivités territoriales, il existe une mosaïque d’outils transfrontaliers – commission intergouvernementale,

Je suis pour ma part convaincu que l’impulsion doit venir de l’échelon intergouvernemental. Les sujets transfrontaliers relèvent des relations entre les deux États. Le Luxembourg n’est pas une collectivité territoriale, c’est un État souverain. C’est C’est en négociant à l’échelle des États que nous pourrons avancer, ainsi que nous l’avons vu dans le domaine fiscal avec les deux avenants à la convention de 2018. C’est bien par des négociations entre les ministres

pourrait constituer le point de départ d’une véritable rénovation de nos méthodes de travail avec notre voisin luxembourgeois. Pour ce faire, cette conférence doit reposer en priorité sur des échanges bilatéraux à l’échelon ministériel, voire entre les deux Premiers ministres. Il n’est en effet pas satisfaisant qu’elle se réduise à une addition de groupes de travail,

120 000 Français travaillent dans le Grand Duché. Nos compatriotes représentent près de la moitié des travailleurs transfrontaliers de ce pays. Ainsi, la France se situe loin devant la Belgique et l’Allemagne, qui sont les deux autres pays à alimenter ce contingent. Cette situation nous rappelle tout d’abord le grand décalage de compétitivité entre la France et le Luxembourg, où le salaire moyen et le PIB par habitant sont nettement plus élevés que chez nous. C’est évidemment et sans aucun doute la principale raison qui explique qu’autant de nos compatriotes aient opté pour ce mode de travail. de travail. Dans la pratique, ce choix est naturellement facilité par l’intégration européenne. Reste que cette dernière ne détermine aucunement le régime d’imposition de ces travailleurs, qui relève du domaine des conventions fiscales bilatérales. La question n’est pas nouvelle la convention bilatérale de 2018 a déjà actualisé les relations fiscales entre nos deux pays au regard des derniers standards de l’OCDE, notamment afin d’éviter les doubles impositions. Cette même convention a déjà été amendée en 2019, afin de mieux prendre en compte la situation des travailleurs transfrontaliers, c’est à dire essentiellement des Français travaillant au Luxembourg. avec le développement du télétravail, les règles classiques déterminant le pays d’imposition se révèlent pour partie caduques. À cet égard, on peut dire qu’il en va des règles fiscales comme de toutes les règles : le développement du télétravail, s’il ne les remet pas en cause, oblige le plus souvent à adapter les règles fondamentales du travail. En l’occurrence, l’avenant de 2019 à la convention fiscale a déjà précisé la règle pour l’imposition des télétravailleurs, en fixant un forfait de 29 jours télétravaillés. En deçà de ce plafond, les travailleurs continuent d’être imposés dans l’État de situation de l’employeur, c’est à dire au Luxembourg. Au delà, la totalité des jours télétravaillés est imposée dans l’État de résidence. Le projet de loi aujourd’hui soumis à l’approbation du Sénat propose de relever ce plafond de 29 à 34 jours, ce qui va dans le bon sens, ainsi que le rapporteur l’a fait remarquer. Ce relèvement présente au moins deux avantages. En premier lieu, il apporte sécurité et confort à tous les travailleurs transfrontaliers qui exercent au Luxembourg un emploi pour lequel le Certes, comme cela a déjà été rappelé, on ne sait pas bien comment l’application de ce plafond sera contrôlée. En tout état de cause, s’il peut y avoir une zone grise, mieux vaut pour les transfrontaliers transfrontaliers qu’elle se situe autour de 34 jours plutôt que de 29 jours. En second lieu, le rehaussement de ce plafond répond à une demande des autorités luxembourgeoises. On comprend bien l’intérêt de celles ci, puisqu’un tel relèvement implique des recettes fiscales supplémentaires. Toutefois, puisqu’il est également clair que des dizaines de milliers de nos compatriotes tirent profit de leur situation de travailleur transfrontalier,

le Luxembourg est un partenaire économique important de notre pays. En 2022, la France reste son troisième fournisseur et son deuxième client. En matière de services, le volume des échanges a atteint 16,3 milliards d’euros

ainsi que d’une clause générale anti abus. Depuis l’adoption de cette convention, le Luxembourg s’est mobilisé en matière de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, et le Grand Duché constitue l’un de nos partenaires essentiels.

En effet, la crise sanitaire a bouleversé l’organisation du travail. Elle a favorisé un recours beaucoup plus fréquent au travail à distance, qui s’effectue parfois depuis un pays différent. ne pouvait pas être pris en compte dans la convention de 2018. Le Luxembourg est particulièrement dépendant de la main d’œuvre transfrontalière, compte tenu de sa superficie et de sa situation géographique : près de 121 000 de 121 000 transfrontaliers Français travaillent au Luxembourg. Dans le détail, le protocole annexé à la convention de 2018 prévoit un forfait de télétravail de 29 jours au cours duquel le contribuable est supposé travailler dans l’autre État. Concrètement, un Français qui télétravaille qui télétravaille en France moins de 29 jours est réputé exercer son emploi au Luxembourg et continue donc d’être imposé dans ce pays. En revanche, s’il dépasse ce seuil, son activité sera imposée dans son État de résidence

et la Belgique ou l’Allemagne, afin de placer les travailleurs transfrontaliers sur un pied d’égalité, quel que soit leur pays d’origine. Si ce régime permet de simplifier la situation des transfrontaliers, il conduit pour la France à une perte fiscale estimée entre 30 millions d’euros et La seconde grande mesure de cet avenant vise à étendre le bénéfice du forfait de télétravail à certains contribuables percevant des rémunérations publiques. La convention de 2018 précise que les rémunérations publiques sont imposées dans l’État de source. Ainsi, un Français travaillant au Luxembourg pour l’ambassade de France est imposé en France. Par exception, la convention stipule que les rémunérations publiques sont imposées dans l’État d’exercice de l’activité lorsque le contribuable est résident de cet État et dispose de sa seule nationalité. Ainsi, un Luxembourgeois qui travaille au Luxembourg pour l’ambassade de France est imposé au Luxembourg. Or le télétravail peut faire basculer un contribuable d’une hypothèse à l’autre. Un Français qui travaille pour la ville de Luxembourg est imposé au Luxembourg en présentiel, mais en France en télétravail. Pour remédier à cette situation, l’avenant prévoit qu’en deçà du seuil de 34 jours de télétravail les revenus sont imposés dans l’État de source, afin d’aligner le régime des personnes employées dans le secteur public sur celui du secteur privé.

à la convention fiscale franco suisse de 1966. Celui ci prévoit un forfait de télétravail à hauteur de 40 % du temps de travail, soit deux jours par semaine, au cours duquel s’applique le principe d’imposition dans l’État d’exercice de l’activité. En contrepartie, l’État qui dispose du droit d’imposer reverse une compensation fiscale à l’État de résidence. Une telle solution pourrait servir de base pour un nouveau régime d’imposition du télétravail transfrontalier avec le Grand Duché du Luxembourg. des travailleurs transfrontaliers reste néanmoins un sujet de préoccupation. Dans l’immense majorité des cas, il s’agit de personnes qui résident en France et travaillent au Luxembourg. Ils sont donc redevables de leur impôt sur le revenu au Luxembourg. Leur présence sur le territoire français se traduit par des dépenses élevées pour les services publics, sans que la France ni les collectivités obtiennent de justes retours fiscaux. Cette situation pose un véritable problème.

l’a indiqué. L’évitement fiscal est d’autant plus condamnable que les entreprises qui optimisent leurs impôts à l’étranger sont souvent de grandes utilisatrices d’infrastructures publiques.

nous examinons aujourd’hui un nouvel avenant à la jeune convention fiscale qui nous lie au Grand Duché du Luxembourg et qui vise à éviter la double imposition ainsi qu’à prévenir l’évasion et la fraude fiscales. concerne principalement les travailleurs transfrontaliers qui occupent des postes dans lesquels le télétravail est possible., la convention de 2018 semble presque visionnaire : elle visait à organiser les conditions de la pratique du télétravail, deux ans avant la pandémie de covid de covid 19. La mise en œuvre du télétravail et son développement sont plus que nécessaires dans cette zone géographique où les transports publics sont malheureusement lacunaires et où les axes routiers sont totalement saturés.

d’une convention pérenne. Le Gouvernement doit y travailler dès maintenant. En effet, un nouvel avenant, à la durée réduite, ne saurait offrir un cadre sécurisé ni aux travailleurs, ni aux entreprises, ni à l’administration fiscale française.

De manière globale, rappelons notre attachement à l’évaluation dans le temps des conséquences économiques et budgétaires de ces négociations fiscales internationales, au traitement égalitaire de tous les travailleurs transfrontaliers,

un projet politique. Cet accommodement représente une perte de recettes fiscales pour la France de 40 millions à 70 millions d’euros. Nous parlons d’un avenant à une convention fiscale qui se refuse à traiter les problématiques soulevées par les LuxLeaks et les OpenLux. La

discrétionnaires de l’administration fiscale luxembourgeoise particulièrement avantageuses ? Où en sommes nous des 100 milliards d’actifs de Français et Françaises logés dans ce paradis fiscal ? En 2020, à la cinquième place du podium des profits dissimulés, nous retrouvons, derrière les Îles Vierges britanniques, le Luxembourg, avec 48,8 milliards Nous avons appris ce lundi que le gouvernement français va prolonger le moratoire concernant l’application de la convention fiscale pour les foyers fiscaux aux revenus mixtes. C’est la troisième année consécutive ! Du provisoire qui dure ! Une raison de plus de réviser cette convention. Mais cette révision ne viendra pas aujourd’hui, et je le regrette. J’ai conscience que mon département, la Meurthe et Moselle, compte parmi les principaux pourvoyeurs de travailleurs du Luxembourg. Le télétravail, qui concerne 9 % d’entre eux, apparaît comme une bénédiction pour certains, une bonne moitié selon les statistiques disponibles. La perte de recettes fiscales est très mal évaluée. Elle avoisinerait les 60 millions d’euros. Être imposé au Luxembourg quand on travaille en France est décidément intéressant d’un point de vue fiscal. Dans la limite de trente quatre jours désormais… Par ailleurs, je crains que la clause de revoyure prévue par le présent accord sous l’impulsion du Grand Duché ne nous conduise à encore accroître le nombre de jours exemptés d’imposition en France. La pression du patronat luxembourgeois se fait forte, si bien qu’il réclame désormais jours après avoir gagné que, sous 50 % du temps de travail, les travailleurs transfrontaliers cotisent dans leurs pays de salariat. est que le Luxembourg ne peut pas se passer de nos travailleuses et travailleurs, dont les cadres frontaliers surdiplômés qui vont chercher un eldorado financier là où le PIB par habitant est trois fois supérieur à celui de notre pays. Les salaires ne connaissent pas la crise de l’autre côté de la frontière. Les ambitions du patronat ne doivent pas être satisfaites, et cet avenant, transitoire, risque de se faire au détriment des finances et de l’organisation des services publics français. La situation est grave en Meurthe et Moselle. Les services publics accueillent, transportent, soignent, nourrissent tous les citoyens. Le débat sur la contribution légitime du Luxembourg au financement des services publics assumés par les collectivités territoriales n’est pas traité à ce jour. C’est un angle mort, un débat politique que d’aucuns refusent d’assumer : la désorganisation des cantines, l’afflux d’habitants, les demandes d’infrastructures liées au télétravail ; je pense par exemple aux espaces de travail de travail partagés, aux installations, aux raccordements à la fibre, etc. Qui doit assumer ces coûts ? La question de la contribution du Grand Duché doit être posée, et je la pose résolument. Je me tiens aux côtés des collectivités qui subissent la désorganisation du travail transfrontalier sans bénéficier de retombées. Plus qu’un effort financier, nous attendons une répartition des efforts et des coûts, afin que les travailleuses et travailleurs transfrontaliers soient également des citoyennes et des citoyens français. Et pas des citoyennes et des citoyens uniquement de passage, mais avec un destin lié à la communauté nationale. Nous voterons contre

chers collègues, en 2018, lorsque la nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg a été signée, 90 000 Français se rendaient chaque jour au Luxembourg pour travailler. si c’est 121 000 ou 122 000 –, et leur nombre pourrait doubler d’ici à 2050, un chiffre d’autant plus considérable si on le rapporte aux 660 000 habitants que compte le Luxembourg. Le dynamisme de cette relation franco luxembourgeoise exige de revoir à intervalles réguliers la copie initiale, pour mieux l’adapter aux réalités de la vie quotidienne des travailleurs frontaliers. C’est ainsi le troisième accord en cinq ans sur les relations fiscales entre nos deux pays. Celui ci a pour objet de porter à trente quatre jours le forfait de télétravail des frontaliers employés dans une entreprise ou une administration de l’autre État : trente quatre jours télétravaillés, mais considérés et imposés comme s’ils avaient été effectués dans l’État de l’employeur. Cette disposition s’applique sur les revenus perçus depuis le 1 janvier 2023 et jusqu’à la définition d’une solution que nous espérons pérenne. La crise de la covid 19 a en effet créé un besoin soudain de renforcer le télétravail. Dans un territoire où la mobilité est un enjeu majeur, cette question est loin d’être anodine. Aujourd’hui, l’engorgement est tel, sur les routes et dans les trains, qu’une telle mesure revêt une dimension primordiale pour l’environnement et la santé au travail. Au mois de décembre dernier, un avenant relatif aux transports transfrontaliers, avec 440 millions d’euros investis dans le ferroviaire. Malgré une mobilisation inédite de l’État et des collectivités, les 24 000 places de train prévues en 2030 ne régleront pas le problème à elles seules. Il est donc naturel que cet avenant relatif au télétravail ait soulevé de fortes attentes. Il offre une perspective sécurisante, mais – je l’ai indiqué – de court terme, puisqu’il faudra dès la fin de l’année sceller un nouvel accord entre les autorités des deux pays, ce qui permettra peut être d’aller plus loin. Je l’appelle de mes vœux, comme bon nombre de mes concitoyens. Une rencontre est déjà prévue pour déterminer les conditions qui s’appliqueront à compter de 2025, avec un nouvel avenant à venir. Être voisin du Luxembourg est une chance pour les 120 000 Français qui y ont trouvé un travail. Mais ce sont aussi des spécificités que nous avons à intégrer dans nos politiques publiques, et les forces vives du territoire s’y emploient sans relâche. Je profite de l’occasion pour saluer le travail collectif engagé par les acteurs locaux et l’État, ainsi que les propositions concrètes qui en émanent en prévision de la future commission intergouvernementale (CIG). Mais j’insiste, monsieur le ministre ministre : pour parvenir à l’émergence d’un véritable bassin de vie transfrontalier qui parle à nos concitoyens, le Gouvernement doit s’engager plus avant dans nos relations bilatérales, notamment avec la création d’un comité interministériel transfrontalier.

Monsieur le ministre, je relaie la voix des élus du territoire, qui comptent sur l’appui du Gouvernement pour défendre les propositions concrètes que nous souhaitons voir figurer à l’ordre du jour de la future CIG. À quelques mois des élections européennes, des avancées sur un futur ou probable

Au rythme de l’évolution que connaît la situation, ce ne sera sans doute pas la dernière. « Bien qu’étant de nature fiscale, l’avenant à la convention présentée devant le Sénat est intimement lié à celui sur le renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers, examiné au mois En effet, chaque avenant vise à accompagner le mouvement qui pousse inexorablement nos concitoyens de Moselle et de Meurthe et Moselle à travailler de l’autre côté de la frontière. Au dernier trimestre 2022, plus de la moitié des salariés transfrontaliers que comptait le Luxembourg étaient des résidents français. En tant que Mosellane, je vois ces accords comme une véritable chance pour notre territoire. Ainsi, l’avenant qui nous est présenté vise à améliorer les conditions de vie de nos transfrontaliers, en étendant la durée du forfait de télétravail de vingt neuf Concrètement, en dessous de ce seuil, le contribuable est réputé exercer son activité dans l’État de son employeur, en l’occurrence le Luxembourg, et y être imposé. Demande récurrente et évolution très attendue par nos concitoyens, une telle mesure permettra naturellement une plus grande flexibilité de nos travailleurs. techniquement un travailleur frontalier d’obtenir plus de vingt neuf jours de télétravail actuellement, la multiplication des obligations déclaratives pour l’employeur constitue, bien souvent, un frein administratif pour les entreprises. En conséquence, celles ci cherchent naturellement à limiter l’octroi de télétravail. De même, l’extension de la mesure à certains contribuables percevant des rémunérations publiques est une mesure de justice fiscale. En effet, elle permettra de mettre un terme à une différence de traitement injustifiée et de rendre ainsi plus attractif l’exercice de fonctions publiques sur le territoire du Grand Duché. Enfin – il faut le noter –, cette mesure devrait entraîner un cercle vertueux, qui réduirait par la même occasion les interminables congestions de nos axes routiers et ferroviaires. « Si cette solution est à saluer, elle ne peut néanmoins pas être totalement satisfaisante, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, tout accord international implique des concessions réciproques. « Dans le cas présent, l’État français renoncera de fait à un gain fiscal estimé entre 30 millions et 60 millions d’euros en fonction du nombre de salariés qui bénéficieront du dispositif. telle perte pourrait être en partie compensée par des recettes de TVA supplémentaires, grâce à la consommation de nos travailleurs restés sur le territoire français. « Néanmoins, cette hypothèse n’est absolument pas documentée : l’absence de contrôle spécifique des déclarations de télétravail rend le chiffrage de ces recettes quasiment impossible. De plus, cette solution sera par nature temporaire. En effet, la clause de revoyure prévue par la convention impliquera nécessairement une nouvelle négociation sur la question d’ici à la fin de l’année 2024. Cela modifiera à nouveau l’équilibre fiscal recherché. Il serait souhaitable que nos relations transfrontalières avec le Grand Duché puissent s’inspirer à l’avenir de celles que nous entretenons avec d’autres pays frontaliers. Prenons l’exemple de la Suisse, où ces relations sont fondées sur le principe d’une compensation financière aux départements limitrophes. « L’entretien de nos infrastructures de transport a un coût particulièrement élevé pour les collectivités frontalières, qui ne voient pas toujours le bénéfice des échanges avec nos voisins. telle compensation serait une mesure juste, car elle viendrait contrebalancer l’imposition exclusive des revenus au Grand Duché et permettrait également à nos collectivités territoriales d’amortir partiellement le coût de la mobilité de nos concitoyens. » La parole

ont un certain nombre de facilités, que nous avons d’ailleurs renforcées dans un texte examiné très récemment par votre assemblée. Je souhaite que la CIG puisse se saisir de cette question. Cela ne me paraît pas insurmontable dans la mesure où les deux pays reconnaissent déjà à leurs élus un certain nombre de droits.

le financement de projets d’infrastructures routières et ferroviaires. Notre horizon est d’aboutir non pas à un financement, mais peut être à une forme de pérennisation de ce type de financement.

L’existence au Luxembourg de 55 000 sociétés offshore gérant des actifs dont la valeur atteignait la somme vertigineuse de 6 500 milliards d’euros

Quel état des lieux peut être fait ? Quels montants ont pu être recouvrés ? Les sociétés offshore révélées sont elles toujours actives ? Quelle a été la qualité de la coopération entre les autorités luxembourgeoises et les autorités françaises ?

D’ailleurs, venant de la même région et du même département, je n’ai pas entendu de volonté unanime… En revanche, j’ai bien entendu

convention ? Tout simplement répondre à l’attente généralisée des travailleurs frontaliers pour sécuriser leurs relations fiscales avec le Luxembourg.

après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, avec 126 conventions en vigueur, la France dispose d’un des réseaux de conventions fiscales les plus étendus au monde. Cela répond à un double objectif : d’une part, accompagner le développement de nos entreprises à l’étranger en sécurisant d’un point de vue fiscal leurs opérations et en prévenant la double imposition de nos ressortissants expatriés ; d’autre part, comme l’indique l’intitulé de la convention soumise à votre approbation, prévenir l’évasion. L’action bilatérale de la France va de pair avec notre activisme multilatéral en matière d’harmonisation de la fiscalité ou de transparence. C’est précisément pour répondre à ce double objectif que le Gouvernement a souhaité conclure la présente convention avec la Moldavie, signée le 15 juin 2022. La France et la Moldavie ne sont actuellement liées par aucune convention fiscale depuis que la Moldavie a dénoncé, en 1998, l’accord en vigueur entre la France et l’Union soviétique du 4 octobre 1985, qui s’appliquait jusqu’alors. Il résulte de cette situation que nos deux États appliquent concurremment leur droit interne en matière fiscale, ce qui crée de l’insécurité juridique pour les contribuables davantage susceptibles de se retrouver dans des situations de double imposition. Nos deux pays sont également dénués de tout cadre bilatéral de coopération en matière fiscale. Un projet de convention fiscale avait été signé en 2006, mais la procédure d’approbation du texte a été interrompue du côté français à la suite de l’introduction en Moldavie d’un taux nul d’impôt sur les sociétés. En l’absence de nécessité de prévenir la double imposition de nos entreprises, le projet avait été stoppé, conformément à la politique conventionnelle française. Face aux récentes évolutions moldaves, à savoir la réintroduction d’un impôt sur les sociétés son adhésion au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’OCDE, le projet a pu reprendre. La France et la Moldavie ont ainsi pu entamer la négociation d’une convention fiscale à l’été 2019 sur la base d’un projet de texte soumis par les autorités françaises. Les négociations se sont poursuivies en 2020 et 2021. Dans le cadre de ces négociations, la France a obtenu plusieurs concessions des autorités moldaves en faveur de ses intérêts. concernent pour les plus significatives, d’une part, la limitation des retenues à la source en Moldavie sur les intérêts et redevances de 12 % à, respectivement, 5 % et 6 %, et, d’autre part, le renoncement de la Moldavie à taxer nos prestataires de services de manière plus aisée que les autres types d’entreprises.

Plus précisément, la convention comprend une clause anti abus générale, qui permettra de refuser l’application de la convention lorsqu’un montage ou une transaction sont clairement abusifs. Elle comporte également des dispositions de coopération administrative en matière fiscale, notamment sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts et l’échange de renseignements. Par ailleurs, elle contient de nombreuses stipulations conformes à notre politique conventionnelle, s’agissant de la taxation du trafic international ou du régime d’imposition des revenus des mannequins, artistes et sportifs. De même, les volontaires internationaux en entreprise (VIE) en Moldavie bénéficieront d’un traitement favorable.

France figure au quatrième rang. Près de 240 entreprises françaises, dont les groupes Lactalis, Orange ou Lafarge, y sont déjà implantés, et d’autres ont déjà indiqué qu’elles souhaitaient s’y établir. Une mission conduite par le Medef international est d’ailleurs prévue en Moldavie pour le printemps 2024 afin d’accompagner les entreprises intéressées. Ce cadre juridique clair et prévisible créera un climat propice aux investisseurs, aux entreprises et à la multiplication des échanges commerciaux. Ceux ci ont atteint

Cette convention participe en outre au renforcement de la relation bilatérale, en même temps qu’elle s’inscrit dans la politique de soutien de la France à la trajectoire européenne de la Moldavie. Le gouvernement de ce pays conduit un programme ambitieux en matière de gouvernance et de lutte anticorruption, dans un contexte difficile. La poursuite du conflit en Ukraine a des effets particulièrement déstabilisateurs pour la Moldavie, dont une partie du territoire est de surcroît occupée depuis plus de trente ans par l’armée russe. La présente convention a d’ailleurs été signée à l’occasion de la première visite d’État d’un président de la République française en République de Moldavie depuis la proclamation de l’indépendance de ce pays, il y a trente La visite de la Présidente de la République de Moldavie en France, la semaine dernière, à l’occasion de laquelle les deux chefs d’État ont signé un accord de défense et une feuille de route économique bilatérale, illustre le dynamisme de notre relation bilatérale avec ce pays, par ailleurs notoirement francophile et francophone. La présente convention s’inscrit directement dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route économique bilatérale, puisqu’elle instaurera le cadre juridique fiscal bilatéral de référence pour les investisseurs et opérateurs économiques. Cette convention, soumise à votre approbation, est donc une manifestation très concrète de notre souhait d’approfondir nos relations économiques avec la Moldavie.

le 15 juin 2022 en Moldavie, ce texte a été ratifié le mois suivant par le Parlement moldave, mais il a fallu attendre le début de cette année pour que l’Assemblée nationale

accompagne dorénavant le développement de la Moldavie, puisque l’Agence française de développement (AFD) y possède désormais une antenne et mène des programmes d’accompagnement et de soutien. La convention fiscale

Nous avons choisi, pour ce qui concerne la France, la méthode dite de l’imputation, qui permet d’imputer par crédit d’impôt d’éventuelles impositions moldaves.

je pense, ce qui est une très bonne chose. Ce texte sécurisera la situation des particuliers comme des entreprises par un cadre clair d’élimination des doubles impositions. Contrairement à des conventions fiscales récentes que notre commission a eu l’occasion d’examiner

En dehors des considérations fiscales et économiques, l’entrée en vigueur de cette convention fiscale bilatérale, dans le contexte géopolitique complexe que nous connaissons, est de nature à encourager la Moldavie dans sa démarche

la suspension du dernier accord fiscal entre nos deux pays, en 1998, lorsque la Moldavie dénonça l’accord entre la France et l’Union soviétique, qui datait de 1985 et s’appliquait encore.

S’il y a peu de ressortissants français en Moldavie, les entreprises françaises sont, elles, toujours plus nombreuses à y être implantées, et leur part de marché connaît une croissance de près de 15 % chaque année depuis quelque temps. Ce nouvel accord constitue donc une bonne nouvelle,

assemblée. Les études d’impact, comme le suivi adoption, sont généralement insuffisantes, ce qui se traduit par une absence de vision et de communication d’ensemble au Parlement, que nous ne pouvons que regretter.

par la Moldavie d’un impôt sur les sociétés et son adhésion au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’OCDE qui ont permis de relancer le processus en 2019.

où une grande partie des élèves du secondaire apprennent notre langue. L’Alliance française de Moldavie est l’une des plus importantes d’Europe. Politiquement, elle a engagé un virage très important depuis l’élection de Maia Sandu à la présidence. Nous devons soutenir cette orientation, tant les défis à relever sont importants dans le contexte géopolitique que nous connaissons actuellement. le défi démocratique, d’abord, dans un pays qui fait l’apprentissage de la démocratie et qui est marqué par une corruption contre laquelle le gouvernement actuel lutte avec détermination.

Il y a le défi du rapprochement avec l’Union européenne, enfin. La Moldavie est devenue candidate à l’adhésion en 2022 et a signé en septembre dernier une lettre d’intention sur la coopération bilatérale en matière de défense

Au lendemain du vote favorable de l’Assemblée nationale, puis du Sénat, au soutien à l’Ukraine, quelques jours après la visite de la présidente moldave à Paris, adopter cette convention

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les conventions fiscales constituent un puissant levier de notre diplomatie économique. Avec plus de 120 conventions signées, la France dispose du réseau le plus étendu Renforcer ce réseau, c’est renforcer notre influence dans le monde. C’est particulièrement vrai avec la Moldavie, dont l’histoire, la géographie et l’actualité confèrent à cette convention une coloration particulière. C’est d’abord une question d’histoire. Voilà près de quatre décennies que plus aucune convention fiscale ne lie nos deux pays. En effet, le 4 octobre 1985, la Moldavie a décidé de dénoncer la convention franco soviétique qui régissait encore les relations entre nos deux pays sur le plan fiscal. En 2006, puis en 2012, des tentatives pour établir une convention bilatérale entre la France et la Moldavie ont échoué. Les choses se sont débloquées en 2019 : un accord a été trouvé pour aligner nos relations fiscales sur les derniers standards de l’OCDE en la matière. C’est un signal très positif de la part de la Moldavie, qui a signé par ailleurs plusieurs autres conventions de même teneur avec d’autres pays européens. Depuis l’élection de Maia Sandu à la présidence en 2020, la Moldavie n’a cessé de renforcer ses liens avec l’Occident. Elle fait désormais partie des pays officiellement candidats à l’intégration à l’Union européenne. Bien sûr, il lui reste beaucoup de chemin à parcourir pour espérer intégrer un jour l’Union. Mais cette volonté politique démontre une inclination vers l’Occident. Nous aurions tort de la décevoir. Car l’avenir de Moldavie tient aussi à sa géographie : coincée entre la Roumanie et l’Ukraine, son sort dépend pour une large part de ce qui se joue actuellement en Ukraine. Une grande majorité des Moldaves refusent que leur pays vive sous la férule de Vladimir Poutine. À cet égard, la situation en Transnistrie, où les séparatistes œuvrent au rapprochement avec la Russie, est un facteur de déstabilisation géopolitique, tant pour la Moldavie que pour l’Europe. Le rapporteur du projet de loi a d’ailleurs précisé, en commission des finances, que la convention fiscale ne s’appliquerait pas à la Transnistrie, et ce jusqu’à son plein retour sous la souveraineté moldave.

qui est à la fois un outil diplomatique à la main de la France et un pas de plus vers l’Union européenne pour la Moldavie. J’espère que cette convention pourra être rapidement adoptée. En effet, le rythme de la diplomatie tranche parfois avec celui de la politique. Je rappelle ainsi que les négociations ont débuté en 2019 et que la convention n’a été signée qu’en juin 2022. Près de six mois après l’adoption de ce projet de loi par l’Assemblée nationale, il est grand temps que le Sénat adopte également ce texte, pour envoyer un signal fort aux autorités moldaves.

le projet de loi que nous examinons aujourd’hui revêt, au delà des considérations strictement fiscales, une importance géoéconomique et géostratégique majeure, pour la France comme pour la Moldavie. Je me réjouis que cette importance soit enfin reconnue. L’objectif d’une convention fiscale est avant tout d’éviter la double imposition, que ce soit pour les personnes morales ou physiques. Lors de ma visite en Moldavie, en septembre 2018, la France était, avec la Suède, l’un des deux seuls États de l’Union européenne à ne pas avoir de convention fiscale avec la République de Moldavie.

Nous étions convenus que la signature d’une convention fiscale serait ma priorité d’action pour ce pays, afin de favoriser le développement de nos échanges commerciaux. Je remercie Véronique Guillotin, présidente du groupe interparlementaire d’amitié France Moldavie, d’avoir toujours soutenu nos efforts collectifs. Sitôt revenu de Chisinau, j’avais interpellé le ministre de l’économie et des finances sur une situation ubuesque qui obligeait les entreprises françaises souhaitant faire du commerce avec la Moldavie à passer par l’intermédiaire de filiales dans des pays tiers, en particulier les Pays Bas ou la Roumanie, afin d’éviter le risque de double taxation. Il aura fallu les conséquences de la guerre en Ukraine pour accélérer des négociations que le ministère de l’économie ne jugeait pas prioritaires jusqu’alors. Comme le disait Jean Monnet, les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. À la faveur de la visite du Président de la République, le 15 juin 2022, quatre années d’efforts ont été couronnées par la signature d’une convention fiscale bilatérale entre Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, et son homologue moldave, Nicu Popescu. Comme tous ceux qui ont milité pour la signature de cette convention fiscale, je me réjouis de la conclusion de cet accord, qui était très attendu des investisseurs, comme l’avait alors souligné Mme Colonna. Garantir la sécurité juridique aux acteurs économiques en prévenant la fraude fiscale constitue

au détriment de la sécurité juridique des contribuables, susceptibles de se retrouver doublement imposés, et de la prospérité des investissements et des échanges économiques entre nos deux pays. La présente convention fiscale comporte une définition modernisée de la notion d’établissement stable et une clause générale anti abus, en adéquation avec les nouveaux standards de l’OCDE. Elle prévoit un mécanisme clair d’élimination des doubles impositions, au bénéfice des contribuables, qu’il s’agisse des entreprises ou des particuliers. Bénéfiques pour les contribuables, et en particulier pour les 240 entreprises françaises installées en Moldavie, les termes de cette nouvelle convention fiscale le seront aussi pour le Trésor public français. Compte tenu du niveau nécessairement asymétrique des investissements entre la France et la Moldavie, l’abaissement des taux de retenue à la source applicables aux dividendes, aux intérêts et aux redevances assurera un partage des recettes fiscales plus favorable à nos finances publiques. Toujours au titre de la sauvegarde de nos intérêts, et au vu de l’importance de l’aide publique au développement apportée par la France à la Moldavie, je me félicite que la convention fiscale retienne un principe d’imposition exclusive dans l’État de résidence

un accord gagnant gagnant signifie que la Chine gagne deux fois ! Après l’agression russe en Ukraine, l’action diplomatique de la France a tout de suite consisté à soutenir la République de Moldavie, financièrement à travers la plateforme de soutien à la Moldavie, et plus globalement, dans sa démarche d’adhésion à l’Union européenne. Or, en fixant un cadre propre à dynamiser les échanges commerciaux avec ce pays d’Europe orientale, l’adoption de ce projet de loi et, à travers elle, l’approbation de cette convention fiscale bilatérale feraient plus que combler un vide conventionnel. Elles enverraient un signal fort à destination de ce pays frontalier de l’Ukraine, qui a épousé, depuis 2020 et l’accession au pouvoir de Maia Sandu, les valeurs libérales et proeuropéennes. L’attente est grande en Moldavie, où je suis retourné en mars l’an dernier. Je sais que Benoît Mayrand, conseiller des Français de l’étranger, Emmanuel Skoulios, président de la chambre de commerce France Moldavie, et notre ambassadeur Graham Paul suivent à distance cet épilogue.

cette convention fiscale entre la France et la Moldavie comble un vide assez rare dans nos relations internationales avec les autres États. En effet, la Moldavie, depuis son retrait de la convention fiscale entre la France et l’Union soviétique en 1985, était un des très rares pays à ne pas avoir de convention fiscale avec notre pays. Cette convention va permettre de renforcer nos relations avec ce pays limitrophe de l’Ukraine, menacé par l’impérialisme russe de Vladimir Poutine. Elle représente, dans ce contexte, un jalon important dans le processus d’intégration européenne de ce jeune État, indépendant depuis seulement 1991. En faisant le choix de l’Europe et du rapprochement avec ses États membres, la Moldavie opte pour un alignement sur les valeurs démocratiques, sur les principes de l’État de droit et pour la coopération régionale. Cette aspiration coïncide étroitement avec notre vision d’une Europe unie et solidaire, fondée sur le respect mutuel, la coopération et la justice sociale. La convention négociée par le Gouvernement vise non seulement à simplifier les échanges commerciaux et à faciliter les investissements, mais aussi à renforcer le lien culturel et linguistique qui unit nos deux pays. Nous ne devons pas sous estimer l’importance de la francophonie en Moldavie, où la langue française reste enseignée et appréciée. En cette année où l’Union européenne occupe une place singulière dans le débat public, du fait du renouvellement de ses institutions, cette convention est un signal politique fort de notre engagement à soutenir la Moldavie dans son rapprochement avec l’Union européenne. Elle témoigne de notre volonté de bâtir des ponts, de favoriser les échanges économiques et culturels et de participer activement à la stabilité et au développement de cette région stratégique de l’Europe. Je formulerai deux réserves à ce stade. La première concerne l’ampleur de l’étude d’impact fournie par le Gouvernement, qui, cette fois encore, ne nous éclaire pas réellement sur les conséquences de l’entrée en vigueur de cette convention, notamment sur nos recettes fiscales. Dans le contexte français d’austérité budgétaire, marqué par une course à l’économie et un refus catégorique de mobiliser les leviers fiscaux, cette question ne saurait être éludée. Elle est plus large que le périmètre de cette convention franco moldave. De manière globale, nous avons besoin, monsieur le ministre, d’une évaluation fine, dans le temps, des conséquences économiques et budgétaires des négociations fiscales internationales. La seconde réserve concerne la lutte contre l’évasion fiscale. L’alignement sur les standards internationaux pour prévenir la double imposition et la fraude fiscale ne nous semble pas suffisant. L’évasion fiscale prive les États de ressources cruciales pour le financement des services publics et la lutte contre les inégalités. Nous ne pouvons donc nous satisfaire de mesures symboliques ou superficielles. Le Gouvernement doit mener sans relâche un combat contre la fraude fiscale, dans cette convention spécifiquement, comme

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de convention fiscale est sous tendu par la perspective d’une adhésion de la Moldavie à l’Union européenne. La procédure d’adhésion est menée au pas de charge et a été légitimée soudainement après le

le même jour que la Géorgie et trois jours après l’Ukraine. Le 23 juin, le statut de candidat à l’adhésion est accordé par l’Union européenne. En décembre 2023, les dirigeants de l’Union européenne ont ont décidé d’ouvrir les négociations d’adhésion avec la Moldavie et ont invité le Conseil à adopter le cadre de négociations une fois que les mesures pertinentes auront été prises. L’ambition est de mener des réformes sur l’État de droit et dans le mais également dans le secteur économique et financier afin d’accroître l’intégration de la Moldavie au sein du marché intérieur. L’accord d’association est à cet égard une forme de cheval de Troie libéral pour faire tomber les frontières, au nom d’une mondialisation des échanges.

La fin du régime de Vladimir Voronin, président de 2001 à 2009, est marquée par un regain d’intérêt des bailleurs internationaux. La relance économique passe par une politique de rigueur pour tenir les engagements pris à l’égard du Fonds monétaire international. La Moldavie est sans doute l’un des pays où le poids de l’oligarchie dans la vie politique est le plus important. En 2014, les trois principaux oligarques, Vladimir Filat, Vladimir Plahotniuc et Ilan Sor – le parti Sor a été interdit sur décision de la Cour constitutionnelle le 19 juin 2023 –, ont été accusés d’avoir commis le « À eux trois, ils ont dérobé en 2014 l’équivalent de 12 % du PIB du pays ! Les deux derniers ont été contraints à l’exil. Corruption et argent roi ont sévi. En somme, l’intérêt majeur de nouer une relation fiscale avec la Moldavie est d’envoyer un signal en vue de l’adhésion du pays à l’Union européenne. Notre réseau conventionnel couvrait déjà en 2019, selon la Cour des comptes, 97 % des importations et 98 % des exportations. L’excédent commercial de la France avec ce pays ne représentait que 0,018 % du total de nos exportations, soit 105 millions d’euros en 2022, pour 71 millions d’importations. Nous comptons soixante ressortissants français en Moldavie.

Finalement, toutes ces asymétries et l’ambition de faire de la Moldavie un espace de concurrence élargi ont conduit la France à balayer dans cet accord les volontés moldaves : un établissement stable pour les services numériques, disposition que le Sénat a votée à de nombreuses reprises, sur notre initiative ; des dispositions sur les prix de transfert qui profiteront certes à nos finances publiques, mais permettront de délocaliser tous les bénéfices de Moldavie alors que nos multinationales y créent de la valeur ; des retenues à la source bien plus faibles que celles qui sont pratiquées en Moldavie, notamment sur les dividendes.

une part importante de sa main d’œuvre établie à l’étranger, la Moldavie demeure l’un des pays les plus pauvres d’Europe. Son gouvernement, dirigé depuis la fin de l’année 2020 par la présidente Maia Sandu, a à cœur de faire avancer le pays sur la voie du développement économique et du rapprochement avec l’Union européenne. autorisant l’approbation de la convention fiscale bilatérale que nous examinons aujourd’hui traduit la volonté du pays de converger vers les meilleurs standards internationaux, la prospérité et l’État de droit. La présente convention, cela a été dit, est inspirée du modèle standard, élaboré par l’OCDE, des conventions visant à éliminer les risques de double imposition et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales. L’accord ne s’applique pas à la région séparatiste de Transnistrie. On pourrait également s’interroger sur son application dans la région autonome de Gagaouzie. Cet ensemble de localités situées dans le sud du pays forme un territoire discontinu, moins connu certes, mais qui constitue aussi un sujet de préoccupation.

Elle concerne aussi les biens immobiliers, les transports internationaux ou encore les rémunérations des artistes, des sportifs et des mannequins. Une attention particulière a été accordée à la sécurisation des transferts de données à caractère personnel. Dans le contexte international actuel, cette dimension se révèle particulièrement sensible. L’examen de ce projet de loi d’approbation est aussi pour moi l’occasion de m’exprimer en tant que présidente du groupe d’amitié France Moldavie. L’élection présidentielle qui doit se tenir à l’automne prochain aura des conséquences majeures pour l’avenir de la Moldavie et elle s’accompagnera d’un référendum sur une future adhésion à l’Union européenne. À l’approche de ces rendez vous importants, les tentatives de désinformation, déjà bien présentes dans le pays, risquent de se multiplier. Lors de mes déplacements en juillet 2021 et en mai 2022 dans cet État membre de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), j’avais pu constater les défis restant à relever, mais aussi la volonté des dirigeants moldaves d’y parvenir et d’apporter à la population des résultats concrets. Dans le contexte de la poursuite de la guerre en Ukraine, dont nous avons abondamment discuté hier avec le Premier ministre, on entend aussi parler, depuis le début, de tentatives de déstabilisation de la Moldavie.

En 2022, les États membres de l’Union européenne ont accordé à la Moldavie le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne. Au delà de la perspective de long terme, c’est pour nos partenaires moldaves un moyen en soi de moderniser leurs institutions.

Face à la complexité croissante de notre monde globalisé, l’harmonisation fiscale internationale est impérative pour assurer l’équité et la compétitivité de nos citoyens et de nos entreprises.

lesquelles représentent un frein significatif au développement économique, décourageant l’investissement et la mobilité internationale. L’approbation de cette convention simplifiera ainsi les transactions transfrontalières et aidera nos entreprises à se lancer sur de nouveaux marchés, grâce à une clarté fiscale accrue, qui assurera à nos concitoyens et à nos entreprises l’absence d’une double imposition. La mise en œuvre de cette convention permettra par ailleurs de prévenir les abus, l’évasion et la fraude fiscales, conformément aux standards internationaux les plus récents. Elle intégrera notamment les avancées du projet Beps et les derniers standards de l’OCDE en matière d’échanges de renseignements et de procédure amiable entre autorités compétentes. Ces dispositifs sont particulièrement nécessaires alors que l’on constate une croissance de nos échanges commerciaux avec la Moldavie, qui sont passés de 115 millions d’euros en 2019 à plus de 150 millions d’euros en 2022. L’augmentation de 52 % de nos exportations au cours du premier semestre de 2022 démontre l’intensification des relations commerciales. Cette dynamique positive, bien qu’elle soit encore modeste en valeur absolue, est révélatrice du potentiel du marché moldave pour les entreprises françaises et justifie de définir un cadre fiscal bilatéral. L’importance de cette convention ne se limite pas toutefois à ce cadre fiscal. Elle représente aussi un élément clé pour la relation de confiance que nous entretenons avec la Moldavie et contribuera à renforcer son intégration européenne, alors même qu’elle est désormais candidate à l’adhésion à l’Union européenne. Cette convention sera donc à la fois l’occasion de consolider nos relations économiques, mais aussi de renforcer nos liens culturels, voire politiques. En conclusion, le groupe RDPI votera en faveur de la ratification de cette convention, qui permettra, nous le pensons, une plus grande justice fiscale, stimulera le développement de nos relations économiques et participera à l’intégration de la Moldavie dans l’espace européen. À défaut d’être original, j’ai été bref

est suspendue. La séance est reprise. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023 285 du 19 avril 2023 portant extension et

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd’hui pour l’examen d’un texte d’apparence très technique, mais dont les effets seront très concrets. Son adoption est essentielle pour assurer la pérennité de plusieurs évolutions récentes de notre droit dans les collectivités du Pacifique. En effet, le 19 avril dernier, le Gouvernement a étendu et adapté par ordonnance plusieurs mesures du code de la santé publique, déjà en vigueur dans l’Hexagone et les collectivités d’outre mer, afin qu’elles puissent s’appliquer à nos concitoyens polynésiens, calédoniens, calédoniens, wallisiens et futuniens, en tenant compte, bien sûr, de l’organisation particulière de ces territoires. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 74 1 de notre Constitution, qui prévoit une habilitation permanente d’extension des dispositions de droit commun existantes dans les domaines de compétences de l’État. La contrepartie évidente de cette habilitation permanente est que les ordonnances prises sur ce fondement doivent nécessairement être ratifiées par le Parlement, ma présence devant vous cet après midi et la nécessité d’un projet de loi spécifique. En effet, faute d’une ratification expresse des sénateurs et des députés dans un délai de dix huit mois, l’ordonnance deviendrait caduque de plein droit.

Le premier objet de cette ordonnance était en effet de rattraper un certain retard en matière d’applicabilité des lois de bioéthique et d’intégrer des dispositions adoptées depuis 2012. L’ordonnance d’avril 2023 a ainsi rendu applicables dans les trois collectivités françaises du Pacifique les récentes dispositions du code de la santé publique relatives aux recherches impliquant la personne humaine, qui permettent de préciser les conditions dans lesquelles ces recherches peuvent être menées et de garantir la sécurité et la bonne information du participant. Sont notamment visées les dispositions relatives aux comités de protection des personnes. Ensuite, l’ordonnance étend et adapte aux trois territoires français du Pacifique certaines dispositions de la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer

alors que vous avez adopté, dans cet hémicycle, puis au Congrès il y a dix jours, l’inscription dans notre loi fondamentale de la liberté de recourir à l’IVG. L’unification des règles de recours en la matière vient améliorer et sécuriser l’effectivité du droit des femmes à pleinement disposer de leur corps dans tous les territoires de la République.

Là encore, il s’agit de sécuriser des mesures législatives importantes pour l’accès à la santé et à la prévention, afin qu’elles bénéficient à l’ensemble de nos concitoyens. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je ne doute pas que les objectifs du texte qui vous est soumis ce soir, après son examen attentif par la commission des affaires sociales – je remercie d’ailleurs la rapporteure Marie Do Aeschlimann pour le travail qu’elle a effectué –, trouveront un écho favorable au sein de votre assemblée. le répète, d’assurer la pérennité de mesures utiles et importantes concernant les recherches impliquant la personne humaine ou les délais de recours à l’interruption volontaire de grossesse. C’est pourquoi je vous invite à voter ce texte afin que cela soit chose faite. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la dans cet hémicycle pour examiner le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé. Le premier objet de ce texte était de rendre applicables certains volets des récentes lois de bioéthique en matière de recherche, notamment les dispositions se rapportant aux recherches impliquant la personne humaine (RIPH), afin de préciser les conditions dans lesquelles elles peuvent être menées et de garantir la sécurité et la bonne information du participant. Cela représente parfois une mise à jour de plus de dix ans et permet une adaptation de références aux règlements européens applicables. Cette même ordonnance a également étendu et adapté au territoire des îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française les dispositions relatives à l’allongement des délais de recours à l’interruption volontaire de grossesse et à la suppression du délai minimum de réflexion. D’autres extensions et adaptations concernent certains territoires seulement. Je pense aux compétences des sages femmes en matière de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles, pour les îles Wallis et Futuna, ou à la protection par le secret de la prescription de la contraception aux personnes mineures, pour la Polynésie française. L’ordonnance qu’il nous est aujourd’hui proposé de ratifier a été prise sur le fondement de l’article 74 1 de la Constitution, lequel permet au Gouvernement, dans les collectivités relevant de l’article 74 ou encore en Nouvelle Calédonie, d’étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur dans l’Hexagone. Cette extension du droit commun ne peut intervenir que dans les seules matières qui demeurent de la compétence de l’État, après consultation des assemblées des collectivités. Contrepartie de cette habilitation permanente donnée au Gouvernement, une ordonnance prise sur ce fondement doit nécessairement être ratifiée par le Parlement dans un délai de dix Si la ratification d’une ordonnance apparaît un exercice particulièrement encadré, voire contraint, j’ai pu rappeler en commission la portée politique et, surtout, juridique de ce texte. La première question posée par ce texte est celle du respect du partage des compétences. Il faut d’abord admettre que l’intitulé de l’ordonnance du 19 avril 2023 est trompeur, car, si les « diverses dispositions relatives à la santé » de cette ordonnance figurent au sein du code de la santé publique, elles font en réalité intervenir des compétences qui ne relèvent pas de la santé. Surtout, la compétence santé relève du pays en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, l’État ne demeurant compétent en la matière qu’à Wallis et Futuna. Aussi l’examen de ce texte fait il apparaître que les dispositions de bioéthique en matière de recherches impliquant la personne humaine ressortissent de la compétence recherche, assumée par l’État, et que celles qui sont relatives au délai de recours à l’IVG, considérant les avis du Conseil d’État et les décisions du Conseil constitutionnel, relèvent de la garantie des libertés publiques et, donc, de la compétence de l’État. Aucun empiétement de l’État sur une compétence dévolue n’a été soulevé par les territoires. La deuxième question que nous devons traiter est celle de la pertinence des dispositions au regard des réalités locales. Les auditions de la commission ont été particulièrement instructives, alors que ni l’ordonnance ni son projet de loi de ratification ne font l’objet d’une étude d’impact fournie par le Gouvernement. Je regrette par ailleurs que seul l’avis du congrès de la Nouvelle Calédonie ait été reçu par le Gouvernement. Je me dois également de relayer les regrets des territoires quant aux modalités de leur saisine sur des projets d’ordonnances parfois très techniques – vous l’avez dit, madame la ministre ou sur des matières particulièrement sensibles. En Polynésie française comme en Nouvelle Calédonie, l’actualisation du droit en matière de recherche impliquant la personne humaine était une demande forte, et l’ordonnance vient parachever un travail mené avec les services des collectivités. Il s’agit de permettre l’intégration de patients de ces territoires à des recherches cliniques, alors que certaines pathologies peuvent se présenter de manière différente ou chez des profils de populations distincts de ceux de Pour Wallis et Futuna, l’extension de ces mêmes dispositions a été faite à la demande de l’agence de santé, afin de permettre une intégration théorique de patients, la réalité de l’offre de soins ne permettant pas en vérité de l’envisager. En revanche, l’allongement du délai de recours à l’IVG n’a, lui, été sollicité par aucun des trois territoires. L’ensemble des représentants des collectivités ont d’ailleurs souligné la sensibilité particulière du sujet, dans des territoires où la société est bien plus religieuse que dans l’Hexagone. La difficulté d’accès, invoquée en 2022 pour allonger le délai de recours à l’IVG, me semble, pour ces raisons, encore plus discutable, au vu des spécificités et des particularités de ces territoires français du Pacifique. Cette situation caractérise une adaptation très inaboutie du droit, qu’il me paraît indispensable de souligner. En vérité, le Gouvernement a étendu le délai de recours à quatorze semaines au nom de la compétence de l’État en matière de garantie des libertés publiques, sans se soucier de son application effective, et ce alors que l’organisation des soins et les compétences des professionnels de santé relèvent du pays en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, comme la prise en charge par l’assurance maladie. Des questions concrètes demeurent également sans réponse, qu’il s’agisse de la formation des sages femmes à l’IVG instrumentale, de la disponibilité et de la responsabilité des professionnels de santé pour un acte qui n’est pas sans risque, ou encore de l’accès aux centres pratiquant les IVG dans ces territoires. Pour dire les choses clairement, le Gouvernement s’est donné bonne conscience, sans se préoccuper de l’accessibilité à ce droit. La dernière question posée est naturellement celle de l’adoption ou non du présent projet de loi. Elle appelle une réponse plus délicate que je ne l’anticipais lorsque j’ai commencé à instruire ce texte. Délicate sur la forme, car une ratification d’ordonnance n’offre que peu de marges de modifications. En effet, qu’il s’agisse des dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine ou de l’allongement du délai de recours à l’IVG, l’ordonnance du 19 avril 2023 qu’il nous est demandé de ratifier a déjà changé le droit au moment de sa publication. délicate sur le fond. Comme je l’ai rappelé en commission, je n’étais pas sénatrice lors de l’examen de la dernière loi de bioéthique, et pas davantage lors de l’examen de mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement. Je constate que les dispositions relatives aux recherches sur la personne humaine ont parfois été adoptées dans les mêmes termes par le Sénat et l’Assemblée nationale, ou sans désaccord insurmontable au cours de la navette. Je ne peux pas en dire autant de la loi du 2 mars 2022, que le Sénat a rejetée

Ces motions rappelaient le faible taux – moins de 5 % – d’IVG réalisées en 2017 dans les deux dernières semaines du délai légal, alors fixé à douze semaines. Elles soulignaient aussi que les professionnels de santé eux mêmes considéraient cet acte comme d’autant moins anodin qu’il est pratiqué tardivement. Ces arguments

de toute évaluation du besoin et de la capacité des collectivités à la mettre en œuvre, que cette extension par ordonnance n’était pas vraiment opportune. C’est pourquoi, à défaut d’une validation politique, notre commission des affaires sociales a fait le choix d’une validation juridique. Sous les réserves concrètes que j’ai pu exposer, elle a décidé de prendre acte de l’évolution du droit, ouvrant ainsi la voie à la ratification de l’ordonnance. Je formulerai enfin deux regrets, madame la ministre. Le premier concerne les modalités d’extension, qui ne satisfont pas pleinement aux principes de sécurité juridique et d’accessibilité du droit. Le second tient aux lacunes de ce texte. L’ordonnance que le Gouvernement nous demande de ratifier a été publiée en avril 2023, soit voilà près d’un an. Certaines demandes de modification, jugées tout à fait recevables par les services des ministères de la santé et des outre mer, ont été transmises depuis plusieurs semaines par la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française. Or, alors même que j’avais sollicité l’expertise de ces propositions par le ministère et appelé à leur intégration au stade de la discussion au Sénat, aucun amendement n’est prêt à être discuté en vue de compléter ou de corriger l’ordonnance.

Je terminerai sur une note plus générale concernant les outre mer. Ces territoires sont confrontés à des enjeux très concrets d’accès aux soins, alors que la multi insularité est un sujet de complexité majeur. Nos compatriotes du Pacifique font parfois face à des difficultés insoupçonnées lors de déplacements dans l’Hexagone. Que la compétence concernée relève de l’État ou soit dévolue au « pays », les indicateurs de santé publique sont souvent préoccupants et les pathologies particulières méritent des travaux parlementaires plus poussés

extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé. Je tiens tout d’abord à saluer le travail de Mme la rapporteure Marie Do Aeschlimann. Parmi les dispositions qu’il nous est proposé d’adapter à ces trois territoires ultramarins, certaines permettront de rattraper un retard accumulé depuis plus de dix ans. Ce constat illustre l’urgence de replacer nos outre mer au cœur des dispositifs de santé.

ainsi que par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Elles permettront notamment aux populations ultramarines des trois territoires concernés – c’est déjà le cas pour le reste de nos compatriotes – d’avoir accès à des traitements innovants, notamment en participant à des essais thérapeutiques. En l’état actuel du droit, la Polynésie ne peut pas contribuer à ces RIPH, tandis que les capacités de la Nouvelle Calédonie sont limitées. Qu’il s’agisse de traitements contre le cancer pour des patients en échec thérapeutique ou de recherches spécifiques sur des pathologies régionales telles que les arboviroses, la leptospirose ou le rhumatisme articulaire aigu, l’alignement sur le droit en vigueur est plus que bienvenu.

regretter. Sur la question de l’interruption volontaire de grossesse, l’ordonnance étend les dispositions de la loi du 2 mars 2022, qui a notamment conduit à l’allongement du délai de douze à quatorze semaines de grossesse pour recourir à une IVG. Si les dispositions relatives à la recherche étaient une demande clairement formulée par les trois territoires ultramarins dont il est question, je note que cela n’a pas été le cas sur ce point et qu’aucune remontée particulière des professionnels de santé n’y a été signalée. Je rappelle également que le Sénat s’était opposé à plusieurs reprises à cette mesure. Néanmoins, au regard des avis favorables formulés par les assemblées locales et considérant l’hypothèse non souhaitable de l’existence d’un droit différent pour ces trois territoires, la majorité du groupe Les Républicains ne s’opposera pas à cette extension. Cela ne doit pas en revanche nous détourner d’un objectif particulièrement difficile à atteindre : rendre

Le véritable enjeu pour les territoires ultramarins, dont les professionnels auditionnés ont souligné les difficultés propres, est donc de permettre l’accès à l’IVG à toutes les femmes dans les délais impartis, ce qui est loin d’être toujours le cas. Le fossé entre le droit et son application effective sur cette question sensible doit être une priorité. Enfin, tout comme la commission, je regrette que la transmission des avis par les assemblées locales n’ait pu avoir lieu dans de bonnes conditions. Seul l’avis du congrès de la Nouvelle Calédonie a pu être reçu dans les délais impartis et les collectivités ont insisté sur ces contraintes de temps, incompatibles avec la remise d’un avis approfondi et étayé. Associer Associer convenablement nos territoires ultramarins aux décisions qui les concernent implique de leur en donner les moyens. Cela impose également que la rédaction des ordonnances respecte minutieusement les principes d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, auxquels certaines formulations dérogent, notamment au regard de l’application de la technique du « compteur Lifou » dans le cas de la Nouvelle Calédonie. Pour conclure, la majorité du groupe Les Républicains votera en faveur de ce projet de loi. Dans sa globalité, ce dernier permettra aux trois territoires ultramarins concernés de rattraper le retard en matière de recherche et de santé, ce

je souhaite tout d’abord saluer l’intervention de Mme la rapporteure Marie Do Aeschlimann. Grâce à un véritable travail de pédagogie, elle a su rendre plus claire une procédure plutôt obscure au premier abord. L’ordonnance qu’il nous est demandé de ratifier concerne des dispositions relatives à la santé, même si elle touche en réalité les compétences de la recherche et des libertés publiques. D’apparence, l’article unique de ce projet de loi laisse penser à un texte mineur.

Il est tout simplement juste et évident que tous les Français doivent avoir le droit d’accéder également comme patients à des essais thérapeutiques. Toutefois, je ne peux m’empêcher d’espérer que les possibilités de participer à de tels essais seront réelles pour les habitants de Wallis et Futuna, compte tenu de l’offre de soins L’ordonnance étend aussi les dispositions relatives à l’IVG issues de la loi du 2 mars 2022. Enfin, elle étend à Wallis et Futuna uniquement les compétences des sages femmes en matière de dépistage et de traitement des Cette loi représente désormais le droit en vigueur pour les Français de l’Hexagone ; il serait inacceptable que tous les Français ne disposent pas des mêmes libertés en matière d’IVG.

Notre groupe Les Indépendants votera en faveur de ce projet de loi. Il insiste surtout sur la nécessité de renforcer l’accès effectif aux soins dans ces territoires, dont la situation sanitaire est parfois particulièrement préoccupante. La

L’article unique du projet de loi que nous examinons a pour objet de ratifier l’ordonnance du 19 avril 2023 visant à rendre applicables aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, dans leur version applicable en métropole, les dispositions se rapportant aux recherches impliquant la personne humaine soumises au livre I du titre II du code de la santé publique.

Les femmes de Wallis et Futuna bénéficieront désormais d’un allongement des délais de recours à l’interruption volontaire de grossesse à quatorze semaines.

de leurs compétences en matière de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la Polynésie française, cette ordonnance apporte, outre les mêmes avancées relatives à l’IVG, une meilleure protection par le secret de la prescription de la contraception aux personnes mineures ou encore de nouvelles garanties en matière de données des patients.

Or on connaît parfaitement les difficultés que rencontrent nos structures médicales en Polynésie, comme en métropole d’ailleurs. Décider c’est bien, mais prévoir les moyens adaptés, c’est capital si l’on veut parler sincèrement d’avancées. sur une carte la géographie de ma collectivité et imaginez les délais qui s’imposent pour une intervention médicale lorsque l’atoll est dépourvu de structures et de médecin Enfin, cette ordonnance étend également à la Nouvelle Calédonie les dispositions visant à renforcer le droit à l’avortement par l’allongement

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les écologistes voteront ce projet de loi de ratification. L’extension relative aux recherches humaines était fortement attendue et demandée, notamment en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.

L’extension dans les trois collectivités de la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement est également une bonne nouvelle. En allongeant les délais pour recourir à l’IVG dans ces collectivités d’outre mer, on facilite l’accès des femmes de ces territoires à des centres de santé dédiés dédiés pour réaliser des IVG dans les meilleures conditions sanitaires possible. Les obstacles auxquels ces dernières peuvent être confrontées pour obtenir une IVG dans des délais stricts seront ainsi réduits,

Cependant, que dire de la forme ? Continuerons nous à prendre des ordonnances tous les dix ans afin de transposer les lois votées au Parlement sur tel ou tel sujet, comme ici sur la santé ? Est il normal que ces collectivités d’outre mer aient dû attendre pratiquement douze ans avant de bénéficier des mêmes avancées que dans l’Hexagone en matière de recherches impliquant la personne humaine ? en effet, ces territoires ne pouvaient pas intégrer de patients au sein d’essais thérapeutiques, et donc accéder à des traitements innovants. Peut on évaluer la perte de chance pour les patients polynésiens ou néo calédoniens atteints d’un cancer et en échec thérapeutique sur l’une de ces îles du Pacifique ? La question mérite d’être posée de

Nous devons promouvoir l’égalité de la loi tout en garantissant le respect des spécificités et des aspirations des collectivités d’outre mer. Il faut créer un juste équilibre entre l’universalité des nouveaux droits et la reconnaissance de la diversité des contextes locaux et des règles d’autonomie.

les représentants des collectivités concernées par cette ordonnance ont tous déploré les conditions de leur saisine. Ils n’ont pas pu formuler un avis approfondi ni effectuer une analyse juridique détaillée sur les différentes transpositions. Mais encore, un seul avis a été reçu par le Gouvernement, celui de la Nouvelle Calédonie. Bien que l’Assemblée territoriale de Wallis

le Gouvernement propose la ratification d’une ordonnance publiée le 19 avril 2023, qui prévoyait d’étendre des dispositions relatives à la santé aux territoires dits ultramarins du Pacifique. Je tiens d’abord, comme mes collègues, à critiquer l’usage des ordonnances. Elles constituent un détournement des prérogatives du Parlement et ne permettent pas d’associer les syndicats, les associations, les élus et les parlementaires Alors que nous avons célébré la semaine dernière l’inscription de l’avortement dans la Constitution, ce projet de loi rappelle que les femmes kanakes, les Polynésiennes, les Wallisiennes et les Futuniennes ont dû attendre plusieurs années pour bénéficier des mêmes droits que les autres femmes françaises : huit ans pour la prescription d’une contraception d’urgence aux mineures avec la suppression de la notion de détresse ; trois ans pour l’extension du délai de ans pour la possibilité pour les sages femmes de pratiquer des IVG ; douze ans pour la recherche médicale et les essais cliniques. Le fait que le Gouvernement ait mis autant de temps pour allonger les délais pour avorter – en les

La République doit garantir les mêmes droits aux citoyennes sur l’ensemble de son territoire, y compris lorsqu’il s’agit de la suppression du délai minimum de réflexion pour avorter ou de l’application du secret de la prescription de la contraception aux mineures. Les territoires d’outre mer ne sont pas des territoires de seconde zone. Madame la rapporteure, selon vous les femmes auraient moins recours à l’IVG dans nos territoires en raison de la prévalence de la religion. La religion n’est malheureusement pas un contraceptif : les femmes doivent se cacher davantage pour y avorter. Je voudrais par ailleurs relayer les critiques formulées par mon collègue kanak Robert Wienie Xowie sur le manque de lisibilité, d’intelligibilité et d’accessibilité de l’ordonnance du 19 avril En effet, le Congrès de Nouvelle Calédonie a rendu un avis favorable sur le texte et en a critiqué les risques en matière de sécurité juridique. Le non respect des compteurs qui permettent de transcrire les articles dans leur version applicable dans chaque territoire kanak, a conduit la commission permanente à émettre des réserves quant à cette technique d’extension. En effet, celle ci ne permet pas d’identifier clairement les dispositions qui ont vocation à s’appliquer en Nouvelle Calédonie. Enfin, le Congrès a également alerté l’État sur les risques en matière de sécurité juridique que font peser les renvois aux dispositions européennes applicables sur le territoire national. Or les règlements européens ne sont pas directement applicables dans les pays et territoires d’outre mer. Le Gouvernement ne peut donc pas imposer une modification des règles pour les essais cliniques de médicaments ou pour les dispositifs médicaux en invoquant l’application unilatérale des règlements européens. En conclusion,

Si la République française est indivisible, elle doit toutefois s’adapter à certaines particularités. L’article 74 1 de la Constitution permet ainsi au Gouvernement d’étendre par ordonnance aux territoires ultramarins les dispositions de nature législative en vigueur en métropole. Ces ordonnances doivent cependant être ratifiées dans les dix huit mois sous peine d’être frappées de caducité. C’est sur ce fondement qu’a été prise l’ordonnance du 19 avril 2023. nous déplorons que seul l’avis du Congrès de la Nouvelle Calédonie ait été reçu par le Gouvernement dans le délai imparti. Cela a été rappelé : les conditions de saisine des collectivités ne sont pas satisfaisantes et ne permettent pas toujours de rendre un avis étayé sur le fond ni d’assurer une analyse juridique fine. telles que la recherche impliquant la personne humaine, c’est regrettable. L’un des objectifs de l’ordonnance du 19 avril 2023 était en effet de rattraper un important retard dans la transposition des lois de bioéthique en matière de recherche. Elle a ainsi permis de préciser les conditions dans lesquelles ces recherches peuvent être menées et garantissent la sécurité et la bonne information des participants. Elle a par ailleurs permis d’étendre l’application des règlements européens portant sur les essais cliniques de médicaments, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic. Ces adaptations étaient fortement attendues par les trois collectivités françaises du Pacifique. L’ordonnance qu’il nous est proposé de ratifier vise également à étendre à la Polynésie française des dispositions de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, relatives à la protection par le secret de la prescription de la contraception aux personnes mineures.

et la suppression du délai minimum de réflexion à l’issue de l’entretien psychosocial. Quelques jours après avoir fait entrer l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, nous nous réjouissons bien évidemment de la transcription de ces dispositions. Si la liberté des femmes de recourir à l’IVG est désormais « irréversible », pour reprendre les mots du Président de la République, l’accès à ce droit conquis de haute lutte est toujours fragile. Le recours à l’avortement reste inégal

N’oublions pas qu’il aura fallu attendre vingt six ans pour que la loi Veil soit appliquée en Polynésie française. Comme l’a souligné Mme la rapporteure, l’absence de ratification de l’ordonnance du 19 avril 2023 entraînerait un retour au droit antérieur. C’est la raison pour laquelle le groupe du RDSE apportera bien évidemment son soutien à ce projet de loi. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure – je salue à mon tour la qualité de votre travail –, mes chers collègues,

La République accorde aux citoyens des collectivités du Pacifique les divers régimes auxquels ils aspirent dans la liberté, l’égalité et la fraternité qui les lient tous ensemble. Le texte que nous examinons aujourd’hui procède à la nécessaire ratification de l’ordonnance du 19 avril 2023 qui étend en les adaptant, conformément à l’article 74 1 de la Constitution, des dispositions législatives relatives à la santé à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. Il s’agit tout d’abord de mesures relatives à la recherche impliquant la personne humaine, afin de rattraper le retard pris dans l’application des lois bioéthiques depuis 2012 dans ces territoires. Cette ordonnance permet également l’application de la loi sur l’allongement du délai de recours à l’interruption volontaire de grossesse, passé de douze à quatorze semaines.

Vous l’aurez compris, ces différentes mesures étaient nécessaires pour assurer l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire français et permettre aux habitants de ces collectivités d’accéder à de nouveaux droits déjà assurés en métropole, comme l’allongement du délai de recours à l’IVG.

que la ratification de cette ordonnance doit se faire dans les dix huit mois suivant sa promulgation, sans quoi ces mesures deviennent caduques et l’on retourne au droit antérieur. Voter cette ratification, c’est donc donner de la lisibilité et de la sécurité aux acteurs qui mettent en œuvre ces dispositifs au sein de ces territoires. Voter cette ratification, c’est aussi assurer l’effectivité des droits des personnes à tous les citoyens français. Voter cette ratification, c’est enfin tenir compte des spécificités de chacun de nos territoires. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI soutient ce texte et votera en faveur de la ratification de cette

et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé.

l’application des nouvelles dispositions relatives à la bioéthique et des règlements européens portant sur les essais cliniques de médicaments, les dispositifs médicaux et les méthodes de diagnostic. L’ordonnance rend ensuite applicables à ces territoires les évolutions législatives récentes relatives aux droits des personnes malades, à la santé sexuelle, à l’interruption volontaire de grossesse et à différents produits pharmaceutiques. Les modifications majeures

: allongement du délai de recours à l’IVG de douze à quatorze semaines de grossesse, suppression du délai minimal de réflexion de deux jours pour confirmer sa volonté d’avorter, possibilité de recourir à la téléconsultation pour l’avortement, autorisation accordée aux sages femmes de réaliser des IVG par voie instrumentale dans les établissements de santé ou encore élargissement des compétences des sages femmes en matière de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles chez les partenaires des femmes dans le but d’améliorer le système de santé

Autre disposition positive contenue dans cette ordonnance du 19 avril 2023 : l’application à la Polynésie française de la possibilité offerte à un plus grand nombre de professionnels de santé de déroger à l’obligation de recueillir le consentement de l’autorité parentale quand des situations ou des actions de prévention, de dépistage ou de traitement sont nécessaires pour protéger la santé sexuelle et reproductive des mineurs.